qui grèvent le budget de la sécurité sociale à hauteur de 23 milliards d'euros en 2018 et contribuent à maintenir une partie des travailleurs à de bas niveaux de rémunération et de qualification. Le renforcement des allégements généraux de cotisations patronales sur les salaires modestes prévus par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 conduira à un tassement des salaires en dessous de 1,4 fois pour que les entreprises puissent bénéficier des exonérations sociales. Or 23 milliards d'euros, c'est la somme qui manque à notre enseignement professionnel et à nos universités pour former les ouvriers, cadres et techniciens de demain

créé en 2012, par une suppression définitive des cotisations des entreprises à la branche famille de la sécurité sociale. Or cette

le Gouvernement demande aux plus vulnérables de se serrer la ceinture en ne revalorisant quasiment pas les prestations sociales, en maintenant la hausse de la CSG pour les personnes à la retraite et en supprimant un certain nombre d'aides destinées aux personnes en situation de handicap notamment. Le groupe CRCE estime que les entreprises doivent continuer à participer au financement de l'ensemble du régime de sécurité sociale, dans la mesure où elles sont directement bénéficiaires de prestations familiales. Cette position s'inscrit dans la logique qui a prévalu lors de la création de la sécurité sociale et selon laquelle chacun doit cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Pour ces raisons, nous proposons de rétablir la version antérieure de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait la mise à contribution des entreprises au financement de la branche famille.

Les chambres consulaires assurent elles-mêmes le coût de l'indemnisation chômage de l'ensemble de leurs agents, qu'ils relèvent du droit public ou du droit privé, mais elles ne bénéficieront pas ne bénéficieront pas de l'allégement de charges. Il serait inéquitable qu'elles soient exclues du bénéfice de mesures dont l'application leur permettrait d'employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé

En outre, les chambres consulaires sont les seuls établissements de France sur lesquels pèse la charge de compenser la hausse de la CSG en 2018, faute de dispositif exonérant leurs employeurs des charges correspondantes.

Si le CICE a été créé pour compenser les charges fiscales des entreprises, monsieur le ministre, sa suppression ne doit pas créer de nouvelles iniquités. Il n'est pas acceptable que, parmi les structures qui ne bénéficiaient pas du CICE, certaines aient droit demain à l'allégement de charges, et d'autres

SMIC. Cet amendement vise donc à compenser l'effet négatif de la dégressivité en faisant commencer le bénéfice de l'exonération de charges patronales à 1,3 fois le SMIC pour les associations intermédiaires.

est à M. Philippe Mouiller. Cet amendement, déposé par Michel Raison, a pour objet de clarifier la situation des salariés travaillant en continu, au regard des dispositions législatives relatives à la réduction générale de cotisations et de contributions sociales figurant à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

en Haute-Saône. Créée en 1475, cette entreprise emploie encore 145 salariés, qui sont des ouvriers qualifiés. Son processus de fabrication, reposant sur des coulées, impose un travail en continu dans un environnement très pénible,

alors même qu'ils bénéficient d'une équivalence « temps plein » en vertu de leur contrat de travail. Cette situation a pu conduire à des redressements d'entreprises par les URSSAF. Aussi convient-il de préciser, dans le code de la sécurité sociale, que les salariés travaillant en continu doivent être considérés comme des salariés exerçant à temps complet

en instaurant la possibilité de supprimer les allégements de cotisations pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations légales en la matière.

... Normalement, la loi impose aux entreprises de plus de cinquante salariés de négocier un accord d'entreprise ou d'élaborer un plan d'action en matière d'égalité salariale.

le montant varie selon les circonstances. Or cette pénalité n'est appliquée que dans 0,2 % des cas ... Afin de contraindre réellement les entreprises contrevenantes, nous proposons donc d'instituer une sanction systématique.

En cas de récidive, lorsque l'employeur n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs,

Les entreprises des outre-mer bénéficiaient depuis 2009 d'un dispositif particulier d'exonérations de charges mis en place par la loi pour le développement économique des outre-mer, la LODEOM, plus adapté à leur contexte local que le régime général.

L'étude macroéconomique réalisée par les socioprofessionnels de La Réunion fait ressortir, quant à elle, une perte de 200 millions d'euros. Le rapporteur général du Sénat évalue lui-même le gain pour les finances publiques à 66 millions d'euros.

anonymes ; elles ne sont donc pas confidentielles. Ce manque de transparence est inacceptable et contre-productif. Il laisse à penser qu'il y a des choses à cacher. Madame la ministre, la réforme présentée aujourd'hui n'est pas aboutie elle nécessite encore des discussions et de la concertation. C'est pourquoi je me vois dans l'obligation de vous en demander le report. Cet amendement vise donc à supprimer la réforme des exonérations de charges dans les outre-mer afin de poursuivre les discussions et d'aboutir à un texte accepté par tous les acteurs économiques des territoires concernés, qui pourrait alors être adopté, par exemple dans le PLFSS pour

Magras. Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, cet amendement vise à ajuster le dispositif d'exonérations de cotisations patronales à la situation de Saint-Barthélemy, dans une logique de différenciation territoriale à laquelle, vous le savez, je suis très attaché. Cette adaptation est d'abord nécessaire. En effet, s'il est vrai que l'économie de Saint-Barthélemy affiche des indicateurs plutôt rassurants, une augmentation de la fiscalité sociale ne serait pas sans conséquence et ne se justifierait

En outre, la ventilation des salaires montre que le dispositif issu de la LODEOM assure aux entreprises une réduction du coût du travail plus ajustée à la répartition moyenne de la masse salariale par entreprise, eu égard aux taux d'encadrement. Pour cette raison, le nouveau régime proposé provoquerait, pour les entreprises de Saint-Barthélemy, une augmentation des charges, au contraire de son objectif, qui est de les réduire.

Le coût du travail est, dès lors, un des principaux leviers de compétitivité des entreprises, en particulier de celles du secteur touristique et de sa périphérie, qui doivent, de surcroît, faire face à l'émergence de la concurrence des îles voisines, dont on connaît les écarts en matière de coût du travail. Antérieurement, Saint-Barthélemy ne pouvait évidemment prétendre au CICE, qui était une disposition fiscale. C'est pour tenir compte de la part du coût du travail dans son PIB que le bénéfice des mesures de compétitivité renforcée lui avait été accordé, il y a seulement deux ans. En matière de cotisations et de contributions sociales, Saint-Barthélemy relève du droit commun et, à ce titre, peut légitimement bénéficier des dispositifs de réduction du coût du travail. L'amendement que je vous soumets apparaît donc comme un compromis raisonnable.

euros par heure de charges patronales, contre 2 euros en métropole. Néanmoins, cette mesure ne peut être cumulée avec aucune autre exonération, sauf pour certains publics spécifiques. Le présent amendement

De plus, la planification de l'espace maritime d'ici à 2021 rendra nécessaire la formalisation de l'inclusion de ce secteur dans la politique maritime, ce qui devrait contribuer à son essor. Le nautisme est donc bien un levier de compétitivité pour les économies ultramarines, et, à ce titre, il convient de le rendre éligible aux exonérations prévues pour les secteurs dits « de compétitivité renforcée

je cherche la cohérence ! Aujourd'hui, on nivelle par le bas l'attractivité des salaires. Comment l'expliquer ?

le travail magnifique réalisé par l'ancien sénateur Désiré, le maire de cette commune, qui a refusé la fatalité de la pauvreté, de la misère et du désespoir au sortir de la crise sucrière, faisant de sa ville un pôle tourné vers la mer.

De plus, les entreprises du secteur aérien sous-traitant largement leurs services aéroportuaires, la réduction des charges salariales se répercutera bien entendu en baisse des coûts.

que, par la sous-traitance, le secteur des services d'assistance aéroportuaire fait partie intégrante de l'économie du transport aérien, donc indirectement de celle du tourisme, cet amendement vise à l'intégrer au dispositif prévu, de manière à soutenir la compétitivité de l'ensemble de la filière.

Les professionnels du conseil, les consultants, les bureaux d'études techniques et les experts-comptables ayant une activité légale sur les territoires ultramarins sont encore trop rares. La Réunion compte cent soixante experts-comptables, la Martinique et la Guadeloupe quatre-vingts En Guyane, on observe une corrélation entre la hausse du nombre d'experts-comptables, de onze en 2009 à dix-sept aujourd'hui, et la hausse du taux de déclarations fiscales, passé, dans la même période, de 50 % à 75 %. Néanmoins, ces efforts ne peuvent combler le retard important des territoires ultramarins sur la métropole. S'agissant des bureaux d'études, les difficultés rencontrées dans ces territoires sont comparables. Les secteurs privé et public peinent à faire émerger des projets, à les piloter et à assurer leur suivi effectif. L'État se voit obligé de sortir de ses compétences de droit commun, afin de fournir un soutien en ingénierie aux collectivités locales. Il est donc indispensable qu'un appui soit apporté aux activités de comptabilité, de conseil aux entreprises, d'ingénierie ou d'études techniques. L'amendement n° 295

aux exonérations spécifiques aux départements d'outre-mer prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, dites « exonérations LODEOM ». Le régime de droit commun se traduirait par un renchérissement du coût du travail pour ces employeurs, malgré le renforcement des allégements généraux. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à leur appliquer le barème spécifique aux entreprises de moins de onze salariés et du secteur du bâtiment et des travaux publics : maintien d'une exonération de cotisations totale jusqu'à 1,3 SMIC, puis dégressivité jusqu'à 2 Cependant, la rédaction actuelle ne prend pas suffisamment en compte le transport régional, plus particulièrement les liaisons entre les territoires ultramarins et leur environnement régional direct. Aussi le présent amendement vise-t-il à intégrer cette dimension, afin de mieux considérer la réalité de ces entreprises, mais également d'encourager l'ouverture de nouvelles dessertes entre les outre-mer et leurs voisins régionaux. Pour rappel, l'article 1 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a consacré la stratégie de la Nation en faveur de l'égalité réelle outre-mer, avec le déploiement de politiques de convergence favorisant « l'inclusion des territoires dans leur environnement régional ». À cet égard, l'intégration régionale des outre-mer constitue une priorité à laquelle les entreprises du transport aérien participent activement.

il apparaît très difficile pour les entreprises de différencier leurs effectifs en fonction des destinations, les personnels n'opérant jamais de manière exclusive sur les liaisons visées. Il convient, en outre, de soutenir davantage les entreprises régionales du secteur du transport aérien confrontées à une concurrence internationale extrêmement rude, les compagnies étrangères étant soumises à des règles moins contraignantes que la réglementation européenne, avec, de surcroît, des niveaux de rémunération nettement inférieurs.

aux deux autres dessertes visées par le présent 3°, c'est-à-dire à la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ainsi qu'à la liaison entre les territoires ultramarins eux-mêmes.

l'éligibilité au régime de compétitivité renforcé des secteurs également éligibles à la défiscalisation des investissements productifs, ainsi que les activités de comptabilité- certains d'entre vous l'ont demandé à l'instant -, de conseil aux entreprises et d'ingénierie d'études techniques.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, l'article 8 du PLFSS pour 2019 prévoit de recentrer et de simplifier le dispositif actuel d'exonérations de cotisations figurant à l'article 753-2-1 du code de la sécurité sociale. Sans revenir sur les chiffres qui ont motivé la fusion des il me semble important d'attirer votre attention, madame, monsieur les ministres, sur le fait qu'une application directe de cet article 8 ne prendrait pas en considération le contexte économique spécifique dans lequel évoluent les entreprises de Saint-Martin depuis le passage du cyclone majeur Irma au début du mois de septembre 2017. Pour être tout à fait honnêtes, nous mesurons pleinement le soutien apporté par le Gouvernement dans le cadre de la reconstruction de Saint-Martin, ainsi que de son accompagnement constant depuis le passage des catastrophes naturelles précédemment évoquées.

En outre, la nouvelle définition de la rémunération déterminant le franchissement des seuils, donc l'impact des exonérations de charges qui seront consenties, notamment à Saint-Martin, tient compte d'une base de rémunération annuelle globale brute

de trappe à bas salaires, constituant un frein au développement des entreprises les plus exposées à la concurrence régionale et internationale. C'est pourquoi le présent amendement vise à relever le seuil applicable aux entreprises du nouveau dispositif dit « de compétitivité renforcée Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,3 à 1,6 SMIC, tandis que le point de sortie passerait de 2 à 2,5 SMIC. En adoptant cet amendement, nous redonnerions de l'oxygène à nos entreprises, de l'espoir à nos jeunes diplômés et un avenir aux salariés.

l'on ne peinait pas à en recruter et que, à la limite, en France hexagonale, on pourrait se passer d'exonération sur certains niveaux de salaire. En Martinique, en Guadeloupe, en outre-mer, c'est exactement le contraire, monsieur le ministre. Nous avons besoin de cadres 51 % des personnes inscrites à Pôle emploi sont sans qualification ou très peu qualifiées et ne répondent pas aux besoins de main-d'oeuvre de nos territoires. Aujourd'hui, nous de comptables, de gestionnaires financiers, de professionnels qu'il faut rémunérer à la juste valeur de leurs diplômes et de leurs qualifications. Comment

régional inter-DOM. Nous estimons que la création d'un étage supplémentaire pour distinguer quelques secteurs nuirait à la simplicité, à la lisibilité et à l'efficacité voulues par le Gouvernement.

On propose d'intégrer d'autres catégories professionnelles, comme les particuliers employeurs et les conseils en entreprise, et d'autres secteurs, en particulier l'hébergement des personnes âgées,

exercices pratiques, entreprise par entreprise, secteur par secteur. Voilà de nombreuses semaines que nous rencontrons le milieu économique, et je crois honnêtement que nous allons arriver à une issue la plus juste possible.

pas suffisamment, pris en compte, comme la presse, les transports maritimes, les transports aériens et la communication. Nous avançons aujourd'hui une proposition forte pour la Guyane, qui répond à une demande spécifique de ce territoire. Nous savons que les cas de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont un peu différents, puisqu'il n'y a pas de CICE

Prenons bien en compte ces 500 millions d'euros de CICE pour les territoires d'outre-mer : cela n'est pas banal et n'arrivera pas deux fois. Prenons en compte également le fait que, dans les territoires d'outre-mer,

Pour la Guyane, vous l'avez entendu, la réponse est là. Je pense honnêtement que, avec le travail complémentaire qui va être accompli sur les seuils, la Guyane sortira de cette réforme, au total, dans une

à la hauteur de ce que les territoires d'outre-mer attendent et, surtout, qui réponde aux objectifs du Gouvernement et assure la cohérence entre le cadre national et la prise en compte de la différenciation voulue par le Président de la République dans les territoires d'outre-mer.

la concertation. Si vous estimez que, en quinze jours, vous êtes capable d'apporter des réponses précises à toutes les interrogations qui ont été soulevées, depuis toutes les travées,

l'élégance de ne pas rappeler l'histoire, mais j'ai eu un conseiller budgétaire qui voulait absolument faire passer la réfaction de l'impôt sur les outre-mer. Nous avons tous deux été ministres, vous dans un gouvernement, moi dans un précédent.

J'ai toujours salué votre détermination, votre franchise, votre sincérité et l'art que vous avez d'aller au fond des choses. Je comprends donc que, ce soir, vous soyez dans l'embarras le plus total : comment faire, alors que tout ce qui a été dit sur ces travées participe du bon sens relèvent d'une arithmétique sur laquelle nous avons travaillé et dont nous sommes conscients, parce que nous avons le bonheur- peut-être aussi le malheur, car nous sommes porteurs de leurs doléances -de vivre dans des pays que nous connaissons bien

Je ne suis pas députée : je suis porteuse, ici au Sénat, de la voix de nos territoires, de la voix de mon pays. J'aimerais rentrer dans mon pays avec un certain nombre de réponses consacrant le travail que nous avons accompli. Le débat est ouvert, et l'on n'est pas obligé d'avoir raison sur tout.

non pas des augmentations pléthoriques de budget, mais du bon sens ! C'est le bon sens, en effet, qui réclame que les seuils soient revus, parce que nous avons besoin de recruter des cadres et de faire rentrer des gens dans des pays qui se dépeuplent, comme la Guadeloupe ou la Martinique. Nous avons besoin que les demandes qui ont été exprimées en Guyane avec une grande et légitime virulence soient entendues. Je ne parle même pas de Mayotte. Oui, nous avons besoin d'attendre et d'avoir, main dans la main avec un gouvernement qui nous comprend et ne nous écrase pas,

ces régions ultrapériphériques comme pouvant être des centres, qui ont fait et font rayonner la France dans plusieurs océans. Un vrai travail

Je voudrais faire savoir à mes collègues guyanais que je comprends le bien-fondé de leur approche. Selon eux, la démarche n'étant pas aboutie, il faudrait prolonger d'un an

La Réunion ne ressemble pas à la Guyane, qui ne ressemble pas à Saint-Martin, qui ne ressemble pas à la Guadeloupe ou à la Martinique. Et allez voir encore les territoires du Pacifique ! Ce soir, nous avons simplement fait part

au monde économique de Saint-Martin ce que vous avez déjà compris, monsieur Arnell, à savoir combien il est important d'accepter cette réforme, et que Saint-Martin sera gagnant en bout de course, notamment une fois que l'on aura fini le débat sur la modification des seuils, puisque l'on s'est engagé à une telle mesure. Sur les chiffres, monsieur Patient, vous avez raison de dire que je suis un peu gênée. En effet, je ne peux pas produire

que vous évoquez. Pour mémoire, le système actuel pour les personnes qui bénéficient du CICE s'éteint à 3,5

n'engage pas de dépenses supplémentaires. Oui ! Cette mesure est même en dessous de ce qui existe aujourd'hui. Au contraire, les sommes issues du CICE auraient dû être ajoutées

on est forcé d'avoir des mesures de correction. Justement ! Cela s'appelle l'équité. Cela s'appelle retrouver des marges de manoeuvre pour sortir la tête de l'eau.

mais on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions ? Comment faisons-nous pour nous revoir, et quelles sont les garanties qui nous sont désormais données sur ces quinze jours ?